sur l'ensemble du territoire national doit être atteint respectivement sur le territoire terrestre et au sein de chacune des façades et des bassins maritimes sous souveraineté ou juridiction française.

: La parole est à M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à faire en sorte que les communes soient consultées dans le cadre de la procédure de choix des aires protégées et des espaces sous protection. amendement prévoient notamment qu'une étude d'impact du projet leur soit adressée au plus tard lors de leur saisine pour avis.

fixe un objectif global à l'échelle de l'ensemble du territoire national, hexagonal et ultramarin. De même, les dispositions de cet amendement évoquent 30 % « dont 10 % sous protection forte alors que la stratégie nationale prévoit 10 % de la surface nationale sous protection forte, ce qui est moins ambitieux que l'article 56 dans sa rédaction actuelle. Pour ces raisons, la commission est défavorable à l'amendement n° n° 1434 vise à transformer la dimension programmatique de cet article en lui conférant une valeur impérative. Si l'objectif de 30 % d'aires protégées est en bonne voie d'être atteint à l'échelle nationale-

l'amendement n° 1190 rectifié, j'ai déjà eu l'occasion de souligner que les aires protégées ne sont pas des sanctuaires naturels dont l'homme doit être tenu éloigné. À ce titre, si l'extraction de substances minérales d'intérêt national ne doit pas être écartée, il convient,, de prévoir un régime d'autorisation spécifique et encadré, à tout le moins, par un décret en Conseil d'État et après consultation des gestionnaires des espaces.

que le classement est fait en concertation avec l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble des parties prenantes. Dans la mesure où cette élaboration collégiale permet de procéder à l'évaluation préalable des effets de la mise sous protection des espaces, il n'est pas nécessaire de prévoir expressément

Au-delà de l'échelon régional, où des discussions ont déjà lieu, j'ai souhaité la création de comités de concertation sur la territorialisation

Au sein du réseau des aires protégées, mais aussi de la propriété privée ou publique, il existe des espaces naturels dont le mode de gestion relève de la libre évolution. Par cet amendement, je souhaite introduire un alinéa qui n'enlèvera rien à ce qui figure déjà dans l'article, mais qui ajoutera quelque chose. La plupart de ces espaces en libre évolution ne relèvent d'aucune disposition juridique existante. Or la libre évolution constitue un enjeu à part entière des politiques de conservation en garantissant le maintien des conditions biophysiques des milieux, la spontanéité des processus écologiques, la libre expression des phénomènes de régulation et de résilience et les continuités spatio-temporelles de leurs différentes composantes. La stratégie nationale devrait aussi favoriser ces approches non interventionnistes et garantir ainsi la pluralité des modalités de gestion de la nature, y compris dans une perspective forte d'adaptation au changement climatique. Ces approches sont actuellement déployées avec succès dans plusieurs réseaux, en particulier les réserves biologiques intégrales, certains sites des conservatoires d'espaces naturels et du Conservatoire du littoral et les réserves intégrales de parcs nationaux. Cette libre évolution s'entend bien évidemment avec ou sans activité humaine résiduelle.

environ la moitié de la diversité culturelle du monde : 7 000 langues vivantes, c'est un patrimoine important. Par ailleurs, dans le quotidien de ces peuples autochtones, le lien à leur espace naturel est absolument central. Dans l'histoire,

est l'avis de la commission sur ces trois amendements ? S'agissant de l'amendement n° 426 rectifié l'information préalable des peuples et populations autochtones lors de la création d'aires protégées en dehors du territoire français est déjà une réalité en droit international. Il est donc superflu de l'indiquer dans notre droit national, qui plus est au sein de l'article relatif à la stratégie nationale des aires protégées. Cet amendement à portée déclaratoire n'ajoutant rien à ce que prévoit déjà le droit international, j'émets un avis défavorable. Pour ce qui concerne les amendements en discussion commune n 425

En effet, les financements français consacrés à la création d'aires protégées à l'étranger, notamment dans le cadre de la coopération, respectent les règles internationales de prise en compte du consentement des peuples autochtones, édictées notamment par la Convention sur la diversité biologique. J'aurais pu également vous dire que tous les projets accompagnés par l'Agence française de développement sont soumis à la politique politique de maîtrise des risques environnementaux et sociaux. Ils s'alignent sur les normes du groupe de la Banque mondiale, notamment celles qui sont relatives à l'acquisition des terres, aux restrictions à l'utilisation des terres, à la réinstallation involontaire

Ils sont les plus touchés par notre modèle de civilisation, lequel, décidément, n'est pas un modèle ! Leur vie humaine a autant de valeur que la nôtre.

ainsi libellé : La parole est à Mme Nadège Havet. L'inventaire du patrimoine naturel est un outil essentiel pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées. Il recense l'ensemble des richesses écologiques du territoire national fluvial et marin. Le code de l'environnement prévoit la contribution des maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, à cet inventaire, par la saisie des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalables ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification. Cet amendement vise à expliciter le rôle des maîtres d'ouvrage, en précisant la distinction entre les deux phases de versements de données : la première se situe en amont de l'autorisation et/ou de l'approbation du projet ; la seconde se situe en aval. Il tend également à introduire des modifications rédactionnelles,

la biodiversité et à l'accompagnement du pastoralisme. Nous avons la volonté d'assouplir les obligations d'autofinancement imposées aux communes pour des travaux relatifs aux équipements pastoraux, afin d'améliorer l'équipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les éleveurs, le pastoralisme et le loup, qui a pu revenir sur ces territoires. Cet amendement vise donc à assouplir les règles d'autofinancement qui sont imposées aux communes pour les travaux sur des équipements pastoraux, comme des rénovations ou des constructions de cabanes pastorales. Il permettra de ne plus demander un autofinancement aux communes, qui sont souvent de petite taille et qui avaient des difficultés à réunir ces financements pour des équipements absolument indispensables pour permettre un gardiennage des troupeaux et faciliter la cohabitation de l'homme avec ces espèces protégées.

telle disposition préserve les intérêts économiques du monde pastoral, participe à la survie du loup, espèce protégée, en permettant le financement des équipements pastoraux dans les petites communes n'ayant pas les ressources nécessaires.

Au regard des impacts pour les collectivités et de l'enjeu que représente le droit de préférence pour la politique forestière, en particulier au regard du regroupement, il paraît préférable de mener une réflexion plus générale sur les dispositions à prendre pour répondre aux enjeux de biodiversité,

Si cette mesure contribue à la protection des parcelles forestières par des organismes dont il convient de saluer la qualité de gestion, elle peut également retarder l'objectif de réduire le morcellement de la propriété forestière, qui se caractérise par un

pour laquelle j'étais vraiment attachée à la rédaction de la commission. Je trouverais regrettable que vous reveniez dessus. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

et de mettre à mal le retour à l'équilibre économique d'un secteur touristique sérieusement affecté par la crise liée au covid-19. Sont notamment concernés les commerçants, les professionnels du nautisme, les transporteurs maritimes, les hébergeurs, les hôteliers et les cafetiers. Il convient donc de reporter à 2022 l'application de cet article pour préserver la reprise économique de ces acteurs touristiques. d'un amendement de repli. Le contenu de l'article 56 risque d'empêcher une clientèle de profiter d'espaces naturels protégés après de longs mois de confinement et de mettre à mal le retour à l'équilibre économique d'un secteur touristique sérieusement affecté par la crise

Il n'est pas opportun de différer son entrée en vigueur dans la loi elle-même. Si le maire l'estime nécessaire, ou en cas de circonstances particulières à son territoire, il peut s'abstenir de faire usage de son pouvoir de police. Je le rappelle, ces mesures sont attendues par un grand nombre de maires, dont une partie du territoire communal est concernée par l'hyperfréquentation.

L'article 56 permet de réglementer ou d'interdire l'accès des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales. En l'état, il prévoit que l'autorité compétente pour réglementer ou interdire cet accès est le maire ou bien, lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune, le représentant de l'État dans le département, après avis des maires des communes concernées. Dans certains territoires, le rejet du tourisme va croissant et il est nécessaire d'éviter que la régulation de l'accès aux espaces protégés ne fasse l'objet d'une instrumentalisation ou qu'elle ne mène à des réactions locales exacerbées en l'absence de véritable concertation. Le présent amendement vise ainsi à intégrer au processus de consultation les gestionnaires des espaces protégés. Ils animent le projet de territoire en vue de la protection et de la mise en valeur des sites et peuvent être un établissement public de coopération intercommunale, un parc national ou un parc naturel régional. Cela contribuerait à une prise de décision cohérente entre les différentes autorités sur un territoire. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement tend à soumettre l'exercice du pouvoir de police spéciale du maire en matière d'accès aux espaces protégés à la consultation des collectivités et établissements publics. Cette consultation serait complexe à instaurer et retarderait la mise en oeuvre des mesures de limitation ou d'interdiction, ce qui priverait le maire de la réactivité nécessaire pour prévenir les atteintes causées au milieu par l'hyperfréquentation. La commission est donc défavorable

notamment à limiter des ventes déguisées, qui pourraient être réalisées au moyen de donations fictives. Nous avons veillé, afin de ne pas pénaliser les donations réelles entre vifs, à ce que ce droit de préemption ne s'applique pas à plusieurs cas de donations entre proches, notamment les donations entre ascendants et descendants et les donations entre époux et partenaires d'un Pacs. Il est donc proposé la création d'un nouvel article L. 215-13-1 dans le code de l'urbanisme, à l'instar de ce qui existe déjà pour d'autres droits de préemption, comme celui des

En insérant dans la loi que la présomption d'affectation à l'usage du public des chemins ruraux ne peut pas être renversée par une décision administrative, les chemins ruraux seront mieux protégés uniformément sur le territoire dans leur utilisation publique par les usagers

cette affectation. La commission a souhaité supprimer l'ajout de cette mention par nos collègues députés, cette disposition étant en effet source de complexité pour certaines communes, qui peuvent avoir de bonnes raisons d'aliéner un chemin rural dont elles n'ont plus l'usage et qui engendre des charges de gestion et d'entretien. En audition, l'Association

Cet article tend à donner compétence au maire pour décider de l'entretien des chemins ruraux, alors que cette compétence est actuellement confiée au conseil municipal par l'article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime. Cet amendement vise donc à éviter tout risque de conflit de compétence. Il prévoit également de rattacher les dispositions relatives à la délégation de l'entretien des chemins ruraux

À cet effet, en l'absence d'association syndicale, la commune pourra autoriser une association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public. L'amendement n° 470, présenté par MM. amendement est l'occasion de faire un plaidoyer pour les chemins ruraux, avec toutes les externalités positives qu'ils induisent : maintenir la biodiversité, permettre l'infiltration des eaux, stimuler le tourisme, autoriser les randonnées, accéder aux parcelles agricoles, incarner le patrimoine naturel et historique, ou encore lutter contre l'artificialisation des sols. Tel est le rôle des chemins ruraux C'est pourquoi, mes chers collègues, il faut garder en tête que, lorsque l'on permet l'aliénation parfois abusive de ces chemins, il est nécessaire de s'assurer, avant d'envisager la suppression de l'un d'eux, que celui-ci est réellement désaffecté, ce qui n'est pas toujours le cas. pas toujours le cas. Le présent amendement vise donc, d'une part, à faciliter la délégation aux associations de l'entretien de ces chemins ruraux et, d'autre part, à éviter des aliénations excessives. En somme, il s'agit de préserver ces chemins ruraux dans la mesure du possible. Par ailleurs, je me permets de souligner que les communes ne sont en aucun cas obligées d'entretenir ces chemins. Par conséquent, la préservation de ceux-ci n'engendre aucun coût pour les communes. L'entretien peut être délégué aux associations ou se faire d'une manière tout à fait naturelle. Aussi, pourquoi ne pas essayer de conserver cet élément de notre patrimoine naturel et historique, porteur de tant d'aménités Je vous remercie,

prévoit que la décision d'échange de parcelles modifiant le trajet ou l'emprise de chemin rural ne peut être prise qu'après enquête publique, tout comme les décisions d'aliénation des chemins ruraux.

maire. L'article L. 161-5 du code rural et de la pêche prévoit, dans sa rédaction actuelle, que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. Il n'apparaît pas opportun de transférer cette compétence au conseil municipal. L'avis est donc défavorable.

les chemins ruraux offrent une grande diversité de situations s'agissant de leur relief, de leur taille, mais surtout de leur environnement, par rapport aux lieux d'habitation, propriétés riveraines, espaces naturels ou à leurs relations avec d'autres voies. Cette diversité plaide pour que les communes puissent apprécier chaque situation particulière, afin de garantir une protection effective des chemins ruraux sans que les maires aient à apporter la preuve d'un désintérêt durable du public. Présentée comme une mesure de simplification, la disposition proposée introduit en réalité de la complexité dans la gestion communale des chemins ruraux. Le constat que le désintérêt durable du public résulte d'une cause naturelle et spontanée est plus exigeant que le régime actuel, qui repose sur la cessation de l'affectation à l'usage du public. L'avis est donc défavorable.

d'inutile complexité, d'autant que la formulation de l'article 57 offre la garantie que l'échange respecte la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé, notamment au regard de la biodiversité. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une aliénation, pour laquelle une enquête se justifie pleinement, mais simplement d'un échange de parcelles, souvent contiguës, afin de modifier le tracé du chemin rural. L'avis est défavorable.

rectifié, la rédaction actuelle de l'article 57 permet la délégation à une association non seulement de l'entretien, mais également de la gestion d'un chemin rural à titre gratuit. L'amendement est par conséquent déjà satisfait : j'en demande le retrait ; à défaut, l'avis de la commission

aux propriétaires ou aux entrepreneurs responsables de la dégradation d'un chemin rural. Toutefois, par un renvoi au code de la voirie routière, cette possibilité est limitée à certaines dégradations. Ainsi, seules sont visées les dégradations causées par la circulation de véhicules, ou celles liées aux exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise. Un riverain qui dégraderait un chemin rural en entretenant sa propriété ou lors de travaux qu'il réalise lui-même sur son terrain ne peut pas être soumis à cette contribution spéciale. Le présent amendement prévoit d'élargir la possibilité d'instituer cette contribution, quelle que soit la cause de la dégradation dont serait responsable le particulier ou l'entreprise. Cette disposition doit permettre d'aider les communes, ou les associations syndicales, à remettre en état des chemins ruraux qui jouent un rôle environnemental important, notamment pour la préservation des espèces. Quel afin d'assurer la protection des chemins ruraux sans que la commune ait à prendre en charge systématiquement les réparations. Il est de bonne pratique que la personne responsable de la dégradation soit mise à contribution. L'avis de la commission

ou cessions effectuées par les Safer ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Il paraît logique que l'échange de terrains concernant un chemin rural bénéficie de la même exemption, dans la mesure où cette opération

permet de faciliter les échanges de parcelles. Le motif d'intérêt général justifiant l'absence de perception est caractérisé, dans la mesure où l'opération a pour but d'assurer la desserte du territoire communal. L'avis est favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Ces amendements

une meilleure prise en compte des haies, en prévoyant pour les collectivités un plan de gestion durable des haies en bord de voirie. J'ai déjà largement évoqué les haies lors du débat sur le volet « Se nourrir », et j'ai apprécié d'avoir obtenu un vote favorable sur la préservation des haies et des prairies permanentes. Les haies bocagères sont des leviers majeurs pour atteindre les objectifs de transition climatique dans le secteur agricole, le stockage

Si les agriculteurs sont parfois pointés du doigt pour leur mauvaise gestion des haies et la diminution du linéaire de haies qu'elle entraîne, les collectivités ont également un rôle à jouer dans ce domaine puisqu'elles entretiennent les haies situées en bord de voirie, qui représentent un linéaire non négligeable. En effet, leurs pratiques de gestion des haies sont trop souvent inadaptées : les tailles pratiquées fragilisent les arbres, affaiblissant ainsi leur potentiel de stockage de CO2 et le capital des agriculteurs. Pourtant, de bonnes pratiques en matière de gestion des haies, qui

chaque année, plus de 11 000 kilomètres linéaires de haies disparaissent. C'est un contresens majeur à l'heure de la crise climatique et de l'effondrement de la biodiversité. De bonnes pratiques en matière d'urbanisme, associées à l'instauration d'un dialogue au niveau local, permettent de préserver efficacement le linéaire de haies existant, et de le développer. Des collectivités et des parcs naturels régionaux se sont saisis des bonnes pratiques et mènent un travail qui permet localement une gestion durable du linéaire de haies. Afin d'encourager les collectivités à utiliser ces bonnes pratiques et de reconnaître le rôle majeur de la haie comme outil de stockage du carbone et de préservation de la biodiversité, cet amendement tend à mentionner explicitement les haies dans le code de l'urbanisme, au même niveau que les principes généraux du code, les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCoT). Alors que, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, il nous faudrait doubler le linéaire actuel de haies d'ici à 2050, il est essentiel d'envoyer un signal fort à la fois aux agriculteurs et aux collectivités.

extrêmement consensuel qui ne contraint ni les collectivités ni les agriculteurs, mais incite à des concertations locales, nécessaires, sur ce sujet. Quel de la commission ? Cet amendement prévoit que l'action des collectivités publiques doit chercher à atteindre « le maintien du linéaire de haies existant, la plantation de haies et leur gestion durable ». Il ne me semble pas opportun d'inscrire les haies et leur gestion durable au sein des principes

dans le cadre des PLU ainsi que la protection et la mise en valeur des haies et trames bocagères qui est rendue possible à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit que les éléments du paysage ou secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique puissent être identifiés dans le règlement.

que l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme permet de classer des secteurs au titre des espaces boisés classés, ce qui soumet les coupes éventuelles à la procédure de déclaration préalable. Par ailleurs, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU

année après année, à diminuer en linéaire. Pourtant, la haie bocagère, c'est le couteau suisse de la biodiversité et de la lutte contre le réchauffement climatique. On pourrait faire un plaidoyer qui peut durer très longtemps. À cet endroit, les arbres apportent leur ombre

en train de vivre une baisse drastique de la biodiversité- insectes, oiseaux et autres - ; il est plus que temps de réagir et d'éviter l'effondrement. Nous voterons

annoncées depuis plusieurs mois par l'État, sont censées proposer une « boîte à solutions » juridiques et financières pour traiter le phénomène de l'érosion côtière rencontré par de nombreuses collectivités littorales. Le texte initial présenté en commission prévoyait essentiellement d'autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances, l'intégralité des mesures nécessaires

D'une part, ils réduisent la question de l'adaptation à la problématique de l'érosion littorale, les autres risques naturels étant écartés du projet de loi. D'autre part, leur périmètre d'application est limité à environ 200 communes littorales, considérées comme prioritaires au regard du rythme de recul de leur trait de côte enregistré par l'indicateur national de l'érosion littorale. Non seulement ces articles dissocient le risque de submersion marine et celui d'érosion, en supprimant les plans l'indicateur retenu n'intègre pas les coups de mer, qui peuvent brutalement accélérer le phénomène et rendre son anticipation plus complexe. Nous continuons donc de penser que ces dispositions auraient dû faire l'objet d'un projet de loi en bonne et due forme.

En métropole, les risques d'érosion concernent un quart des côtes et 1,4 million d'habitants résidant dans les secteurs de submersion marine. En outre-mer, les enjeux sont encore plus prégnants. Aujourd'hui, ce projet de loi inquiète les élus du littoral ; je me fais ici la porte-parole de Jean-François Rapin, président de l'Association nationale

au recul du trait de côte. En réalité, ce projet de loi n'est pas l'occasion, pour le Gouvernement, de se saisir du sujet de l'érosion et du recul du trait de côte, mais bien, au contraire, de s'en dessaisir définitivement, en transférant toutes les responsabilités et charges financières aux collectivités. Sur le fond, c'est inacceptable ; sur la forme, cela l'est tout autant. Opérer un transfert de responsabilité et une extension de compétences, au travers d'un amendement gouvernemental, donc sans étude d'impact ni évaluation sincère des coûts, constitue un déni de consultation des collectivités locales et des parlementaires, sur un texte pourtant Madame la ministre, acceptez-le, pour faire face aux défis du changement climatique, de l'érosion et de la montée des eaux sur les littoraux, c'est d'une politique globale, rassemblant l'État, les collectivités, les acteurs économiques et la société civile, que nous avons besoin, non d'un désengagement de l'État, compensé par une hausse de la fiscalité locale. Nous défendons un autre mode d'action partenariale, reposant sur la consultation des communes concernées, sur l'engagement de démarches volontaires, sur la reconnaissance des stratégies locales de gestion du trait de côte et sur l'élaboration d'une convention État-collectivités définissant le plan d'action ainsi que la participation financière des différents acteurs.

La submersion marine menace 1,4 million de résidents français. La Gironde, la Loire-Atlantique, la Seine-Maritime, le Nord et le Pas-de-Calais présentent, à eux seuls, la moitié des résidents permanents vulnérables. Enfin, au moins 850 000 emplois seraient menacés en métropole. Certains jugent les prévisions de l'État dans les plans de prévention trop pessimistes. Pourtant, avec l'actualisation des données scientifiques, l'hypothèse d'une augmentation de 60 centimètres du niveau de la mer d'ici à 2100 semble au contraire plutôt

le dépôt d'un amendement, qui a été déclaré irrecevable, tendant à remplacer le transfert pur et simple des PPRL par une convention de gestion entre l'État et les collectivités intégrant ce plan ainsi que des moyens, notamment la mobilisation des services de l'État pour la cartographie. que soit mis sur pied un réel plan national de prévention des risques, concerté et débattu avec les acteurs concernés, et non arrêté par décret, ainsi que le prévoit cet article.

du trait de côte ; en ce qui concerne la réalisation des projets de recomposition- acquisition du foncier, démolition, renaturation -, les collectivités auront la possibilité de contractualiser avec l'État,

que les collectivités puissent disposer de ressources locales, afin de compléter les crédits nationaux. À ce titre, elles pourront bénéficier de l'appui technique et financier des établissements publics fonciers (EPF), dont les ressources seront adaptées pour réaliser des acquisitions foncières et les travaux nécessaires aux projets de recomposition littorale. Elles pourront également disposer d'une nouvelle ressource fiscale, au travers de l'utilisation de la taxe Gemapi, afin de financer des projets de recomposition littorale. Voilà quelques-uns des exemples que je voulais vous donner pour vous montrer qu'il n'est évidemment pas question de laisser les collectivités seules face à ce problème. Enfin,

En effet, les améliorations prévues à cet article ne portent pas, pour l'instant, sur les plans d'exposition au bruit des aéroports ni sur les servitudes d'utilité publique.

Par ailleurs, dans un souci de simplicité et de lisibilité pour l'ensemble des acteurs, toutes les informations seraient rassemblées dans un seul document- l'état des risques -au lieu d'être dispersées dans plusieurs documents. Cela procède d'une volonté de simplification. Quel est l'avis de la commission Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement me semble s'écarter du périmètre du texte qui nous est soumis. L'exposition d'un bien au bruit d'un aéroport ou sa proximité avec des servitudes d'utilité publique n'ont que peu de lien avec la problématique des risques naturels ou des effets du dérèglement climatique. Je comprends tout à fait la volonté de renforcer l'information des aspirants acquéreurs ou locataires de biens à toutes les problématiques qui pourraient amoindrir la valeur future du bien qu'ils convoitent

à l'Assemblée nationale. En effet, cet alinéa mentionnait l'amélioration du dispositif d'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers « sur les risques naturels et technologiques [ ...] en y intégrant une information sur l'exposition de la zone concernée au recul du trait de côte

Cet amendement vise à lever une ambiguïté quant au périmètre d'application de la réforme relative au recul du trait de côte prévue aux articles 58 B à 58 I.

Afin de clarifier le champ d'application de la réforme relative à l'adaptation face au recul du trait de côte et de ne pas risquer d'alourdir les responsabilités pesant sur les communes littorales, cet amendement tend à réajuster cette définition en ne visant que le risque d'érosion.

travers du prisme de la planification urbaine, qui est entre les mains des collectivités. Or les multiples expériences en cours dans les territoires démontrent souvent que la question de l'érosion côtière n'est qu'une composante de la transition écologique de modèles de développement centrés sur la valorisation touristique des littoraux.

D'après les chiffres du Cerema, à enjeux constants, entre 5 000 et 50 000 logements seront atteints par ce phénomène à l'horizon de 2100, pour une valeur estimée entre 0,8 milliard et 8 milliards d'euros.

jurisprudence et, parallèlement, les moyens des collectivités sont en baisse. La question du financement de la relocalisation reste donc entière. Dès lors, nous continuons de demander la suppression de cet article, afin qu'un véritable dialogue avec toutes les parties prenantes

mais aussi de la remise en cause de l'occupation des sols. Environ 22 % du littoral français est en situation de recul, avec des variations assez fortes d'une zone à l'autre. L'amendement vise à supprimer cet article, afin de permettre de conserver des informations relatives au recul du trait de côte au sein des plans de prévention des risques littoraux. Cela représente un gage de sécurité juridique pour les communes.

adapté a été adopté, cet article est susceptible de rendre plus vulnérables les communes exposées à l'érosion littorale. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer Par la suppression du recul du trait de côte du PPRL, l'article laisse à penser qu'il ne s'agit plus d'un risque, ce qui aurait pour corollaire une responsabilité qui reposerait entièrement et intégralement sur les communes exposées à ce phénomène. Par ailleurs, cela signifierait que l'État que l'État se désengage de cette question, alors qu'il doit jouer son rôle plein et entier en matière de gestion des risques.

Nous avons souhaité conserver cet article, tout en le modifiant de manière à affirmer un principe de subsidiarité et à donner toute leur portée aux stratégies locales. Le dispositif adopté garantit la primauté du PLU sur le PPRL durant la période transitoire entre l'adoption du PLU intégrant les adaptations au recul du trait de côte et la modification du PPRL. Nous avons travaillé sur cette rédaction avec mon collègue Jean-François Rapin, en étroite collaboration avec l'ANEL. Cet article répond donc aux préoccupations des communes littorales. Concrètement, la suppression de cet article 58 C conduirait à faire coexister les règles relatives au trait de côte issues du PLU et celles Les communes décidant de mettre en place une politique de réorganisation spatiale face au risque d'érosion pourront se voir imposer les règles issues du PPRL, lorsque celles-ci sont plus contraignantes. En pratique, si nous supprimons cet article, nous risquons donc d'entraver les décisions des maires et de créer un flou juridique,

intégrée dans les documents d'urbanisme des communes, n'apporte qu'une réponse très réduite aux enjeux territoriaux liés aux risques littoraux. Ce texte annonce une déresponsabilisation de l'État et un transfert de la gestion du trait de côte vers les communes et les EPCI, sans leur donner les moyens techniques et financiers pour y répondre. Par exemple, les territoires qui font face à l'érosion dunaire sont aussi souvent confrontés au phénomène de submersion marine. Ils devraient être accompagnés par les services de l'État pour développer d'autres formes d'occupation de leurs espaces, en accord avec la population, afin de préserver le développement économique, touristique et le maintien des mobilités et du cadre de vie. À l'inverse, les élus de ces territoires voient, au fil des ans, se multiplier textes législatifs ou projets d'ordonnances, et ont le sentiment de devoir assurer toujours plus de contraintes et de responsabilité. La prescription des travaux de démolition d'office par le maire en est un exemple supplémentaire. Les élus et habitants des littoraux ont besoin d'accompagnement technique et financier, pas d'un millefeuille de législation et d'une superposition d'administrations. l'avis de la commission ? L'avis est défavorable sur cet amendement de suppression. Je m'associe au constat formulé par Mme Gosselin, selon lequel la stratégie proposée n'est pas totalement aboutie, en tant qu'elle n'aborde pas la question des risques littoraux dans sa globalité. J'ai, d'ailleurs, eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet : il me semble que ce projet de loi n'est pas le véhicule le plus adapté pour traiter la problématique des littoraux. Concernant le transfert de compétences opéré vers les collectivités territoriales pour la gestion du recul du trait de côte, je partage également le constat de l'absence de moyens techniques et financiers prévus par l'État pour accompagner la réforme. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit en commission un droit d'option au bénéfice des communes littorales. Nous avons travaillé sur cet article en collaboration avec les élus des communes littorales, sein de l'ANEL. Notre objectif a été de doter les collectivités qui le souhaitent d'outils pour s'adapter face au risque d'érosion tout en les laissant libres d'assumer ou non cette compétence de gestion du recul du trait de côte. Je suis donc défavorable à cet amendement de suppression. Quel est l'avis du Gouvernement ? Il me

comme vous le proposez, la cartographie des zonages relatifs au recul du trait de côte revient à refuser aux acquéreurs et aux locataires de bénéficier du principe d'information préventive avant une transaction immobilière. Cela revient également à leur refuser la possibilité de faire le choix d'une installation sur le littoral en connaissance des phénomènes susceptibles d'affecter leur bien.

est à Mme la ministre. Lors des travaux en commission, vous avez généralisé le droit d'option, y compris pour les communes les plus exposées au recul du trait de côte et non couvertes par un plan de prévention des risques littoraux traitant de l'érosion. Or il y a un réel intérêt, pour ces collectivités les plus exposées au phénomène, à se saisir de tous les outils introduits par le présent projet de loi pour faciliter la mise en oeuvre de leur projet de territoire. L'objectif de cet article 58 E est, tout d'abord, de faire en sorte

égard- c'est important -que les collectivités bénéficieront d'accompagnements financiers et en ingénierie, lesquels permettront de faciliter la mise en oeuvre de cette politique publique visant à protéger nos concitoyens des effets du changement climatique.

appui technique et financier des établissements publics fonciers dont les ressources seront adaptées, d'une utilisation de la taxe Gemapi pour financer des projets de recomposition du littoral. Cet amendement vise donc à rétablir, dans certains cas très ciblés, le caractère obligatoire de l'établissement d'un zonage d'exposition au recul de traits de côtes dans les documents d'urbanisme et le délai associé.

des règles d'urbanisme et d'occupation des sols, tels que les prévoit le projet de loi, vont dans le bon sens. Néanmoins, il faut laisser le temps aux communes potentiellement concernées de s'adapter. La commission a procédé à quelques modifications allant dans ce sens en laissant le choix aux communes de mettre en oeuvre ou non la cartographie du recul du trait de côte et les mesures d'adaptation nécessaires en matière d'urbanisme. Notre Notre commission a décidé d'allonger à cinq ans, au lieu de deux ans, le délai laissé aux communes pour intégrer le recul du trait de côtes dans leurs documents d'urbanisme. Madame la ministre, vous l'avez annoncé vous-même, entre des délibérations, des consultations pour trouver des cabinets spécialisés,

de la commission ? Madame la ministre, je ne suis pas favorable à la suppression du droit d'option. Les garanties apportées par le Gouvernement ne m'apparaissent pas suffisantes concernant le financement de la réforme. D'une part, aucun dispositif de financement national n'est prévu pour cette réforme dans le projet de loi, le Gouvernement renvoyant au projet de loi de finances pour 2022 l'instauration d'une dotation financière. L'idée d'une dotation me semble intéressante, car elle permettrait d'introduire un financement fondé sur la solidarité nationale. Toutefois, les montants évoqués, qui s'élèveraient à 20 millions d'euros, sont malheureusement minimes par rapport aux enjeux. Je rappelle que le Cerema chiffrait les coûts liés à l'érosion dans une fourchette de 800 millions à 8 milliards d'euros. Certes, cette estimation prend comme date butoir l'année 2100, mais elle ne tient compte que des dépenses liées au logement. Les coûts liés aux autres infrastructures et équipements qui seront touchés par le recul du trait de côte, tels que les routes, les stations d'épuration ou les équipements touristiques, ne sont pas pris en compte dans ce chiffrage. Au total, le coût de l'adaptation du littoral au recul du trait de côte risque de s'élever à plusieurs milliards d'euros. Il n'est ni responsable ni réaliste de faire reposer ces coûts sur les collectivités. D'autre part, le Gouvernement propose de financer une partie de la réforme grâce à la taxe je suis plus que dubitatif : la taxe Gemapi peine déjà, par son rendement, à couvrir les besoins relatifs à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. Par ailleurs, faire reposer le financement de la réforme sur la taxe Gemapi revient à faire peser une responsabilité politique et financière très forte sur les élus locaux, qui devront justifier de hausses de la fiscalité locale.

en commission, à cinq ans le délai initialement prévu à deux ans, afin de laisser le temps à une ingénierie qualifiée de se mettre en place et de conférer plus de souplesse aux communes littorales. Il me semble que ce délai est satisfaisant ; il conserve la possibilité pour l'organe délibérant de l'autorité compétente d'établir une carte de préfiguration à titre conservatoire au bout de cinq ans en attendant l'adoption du PLU mis à jour. Toutefois, je ne suis pas fermé à l'étude d'un allongement de ce délai à six ans, si vous l'estimez nécessaire. Je m'en remets donc à la sagesse de notre assemblée.

ans -pour la sécurité des personnes. Néanmoins, la rédaction proposée pose des difficultés sur le fond : elle renvoie aux « constructions autorisées en application de l'article L. 121-22-4 » qui sont situées dans la zone exposée à l'érosion à l'horizon de trente alors que cette règle de démolition s'applique exclusivement à la zone exposée au risque d'érosion à l'horizon de trente ans à cent ans, qui est soumise à un régime différent. Je demande le retrait de ces amendements au profit de mon amendement n° 2300 ; à défaut, j'émettrai

souligne l'imprévisibilité de l'érosion et conteste donc l'approche retenue par le Gouvernement. Ces scientifiques dénoncent un projet de loi guidé par la volonté de préservation du budget de l'État plus que par un véritable raisonnement scientifique.

Si l'on fixait cette taxe à son niveau maximal, il faudrait trois cents ans à la communauté de communes Médoc Atlantique pour qu'elle puisse financer l'adaptation nécessaire de la station de Lacanau.

également de l'anxiété au regard de la responsabilité financière qui pèsera sur eux, mais aussi de la responsabilité juridique. Or cet article 58 G instaure un droit de préemption.

Quel sera véritablement le reste à charge de ces communes ? Il risque d'être important. Pour ce qui concerne le régime de responsabilité, il pèserait sur le bénéficiaire qui n'aurait pas exercé son droit de préemption sur un bien dont il sait pertinemment que, du fait de sa situation, il est situé

qui pèserait sur le titulaire du droit de préemption, mais je souhaite rassurer M. Houllegatte sur deux points. D'une part, le dispositif d'information des acquéreurs et locataires a été renforcé en commission de manière à pleinement intégrer la question du recul du trait de côte. Il me semble que cela va également dans le sens de la protection des autorités compétentes en matière d'urbanisme. Si un incident survient sur un bien sur lequel la commune n'a pas exercé son droit de préemption, il me semble- toutes précautions prises -que le propriétaire pourra difficilement engager la responsabilité du maire, puisqu'il aura été informé de l'état des risques en amont de la vente. Il aura donc signé l'acte de vente en connaissance de cause. D'autre part, le droit d'option que nous avons introduit en commission à l'article 58 E, concernant la mise en oeuvre de la réforme relative au recul du trait de côte, me semble apporter des garanties sur ce point. Le droit de préemption ne pourra pas s'appliquer si une commune a choisi de ne pas délimiter sur son territoire les zones exposées au recul du trait de côte. Quel est l'avis du

aux inquiétudes légitimes d'un certain nombre de maires ou de responsables de collectivités qui voient ce qui est en train de se passer et qui se sentent fort dépourvus. Supprimer l'article 58 G reviendrait à limiter les capacités d'intervention des collectivités locales concernées, alors même que nous oeuvrons à apporter des réponses aux questions que vous soulevez, en particulier sur les mécanismes Ainsi, comme j'ai pu le déclarer précédemment, des moyens financiers seront mobilisés pour soutenir et assurer la mise en oeuvre du dispositif. Je veux être très claire : il y a une part de solidarité nationale dans le financement,

apportent aussi leur ingénierie aux collectivités territoriales, en particulier lorsque les opérations sont complexes. En ce sens, ils pourront être délégataires du droit de préemption créé. Pour ce qui

aux Safer de poursuivre efficacement leurs missions sur les territoires littoraux, spécialement la préservation des espaces agricoles et des activités agricoles du littoral. à exclure les biens immobiliers non bâtis ainsi que les bâtiments d'exploitation, au sens de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, du champ d'application du nouveau droit de préemption prévu par l'article 58 G.

n'a pu obtenir d'éléments précis sur l'impact de cette exemption, notamment sur le nombre et la superficie des biens qui seraient ainsi retirés de l'assiette du droit de préemption. Or il paraît indispensable de veiller à ne pas rigidifier le dispositif. Je rappelle que les surfaces agricoles constituent 45 % du territoire des communes littorales. L'adoption de cette mesure risque donc de priver le droit de préemption de son effectivité. D'autre part, nous avons déjà adopté en commission une rédaction aménageant l'exercice du droit de préemption pour les biens agricoles

prévalait sur le droit de préemption des Safer, mais ne l'excluait pas. En effet, le droit de préemption des Safer pourra toujours s'appliquer en second rang pour des biens soumis au droit de préemption relatif au trait de côte, de la même façon que pour les autres droits de préemption du code de l'urbanisme, en particulier le droit de préemption des espaces

Le titulaire de ce nouveau droit de préemption doit avoir le choix. Si les Safer sont associés suffisamment en amont aux projets locaux, l'articulation entre leur rôle et celui des autres acteurs, notamment les EPF, pourra être organisée au regard de l'ensemble des outils disponibles. le sens donné au texte par l'amendement de M. le rapporteur, qui a été adopté en commission : il est précisé que le droit de préemption relatif au trait de côte pourra s'exercer en coopération avec la Safer pour ce type de biens. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

met en évidence que « les agences n'ont pas été dotées de pouvoir de police, comme le sont les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), le Conservatoire du littoral ou l'Office Alors que leur présence sur le terrain leur permet de suivre les nouvelles constructions illicites en temps réel, elles doivent en référer aux DEAL pour dresser les procès-verbaux, circuit qui, compte tenu des moyens dont disposent ces dernières, manque véritablement de réactivité

Filleul. Cet amendement vise à mieux encadrer les cessions de parcelles dans la zone des cinquante pas géométriques. L'État doit veiller à ce que la décote préconisée par le rapport du CGEDD du mois de janvier 2020 relatif aux cinquante pas géométriques en vue des cessions de parcelles, ne donne pas lieu à des abus fonciers et à des enrichissements sans cause. L'achat de parcelles de grande superficie, ensuite revendues par de nouveaux propriétaires à des particuliers ou à des promoteurs immobiliers

de régularisation dans la zone des cinquante pas, d'autant que les communes ou les agences des cinquante pas géométriques, qui disposent d'un droit de préemption sur les terrains en vente dans cette zone, l'exercent rarement du fait de finances dans le rouge. Par ailleurs, l'État doit privilégier une cession au prix du marché réel en fonction des ressources de chaque demandeur ou foyer domicilié sur place, dans une limite impérative de cinq cents mètres carrés de parcelle, afin de lutter contre l'artificialisation effrénée des différents ultramarins des cinquante pas géométriques et de limiter le nombre de foyers exposés aux risques naturels. Quel de cet amendement trouve une articulation avec le projet de loi 3DS, qui sera bientôt examiné par le Sénat. Il s'agit d'encadrer les cessions de parcelles effectuées par les agences des cinquante pas géométriques en Martinique et en Guadeloupe. Je n'y suis pas défavorable

pour acquérir des terrains déclassés du domaine public à leur profit. Pour faciliter leur régularisation, la loi prévoit que ces parcelles puissent être rétrocédées avec une décote. En revanche, imposer une surface maximale pour les cessions, comme cela est proposé, cela est proposé, pourrait constituer un frein à la régularisation et nécessiterait un nouveau découpage parcellaire, au motif que la parcelle est trop importante. Or, en cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien acquis réalisée dans un délai de moins de vingt ans, le taux de décote doit être remboursé à l'État,

leur permettant d'assurer une préservation efficace et vertueuse des domaines des cinquante pas géométriques et de sanctionner les infractions au code de l'environnement qui peuvent y être constatées. Le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) du relatif aux cinquante pas géométriques aux Antilles prévoit qu'« une voie similaire aux compétences de garderie du domaine conférées au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourrait être mise en place par la loi en prévoyant le commissionnement des agents des agences dans des termes analogues

? Cet amendement va dans le sens d'un renforcement de la protection de la zone des cinquante pas géométriques, qui revêt de forts enjeux en termes de protection de l'environnement, de la biodiversité et des paysages, mais aussi d'accès du public au littoral, et de protection face aux risques naturels, puisqu'ils constituent des zones tampons entre terre et mer fortement soumises aux aléas climatiques. Toutefois, ma chère collègue, je m'interroge sur le caractère opérant de la rédaction retenue. Je pense notamment au périmètre d'application qui mentionne les collectivités régies

de la zone des cinquante pas géométriques aux Antilles. Les recommandations de ce rapport ont été formulées à la suite de nombreuses auditions des acteurs locaux et elles constituent une solution globale à la gestion de ces espaces littoraux. Les collectivités territoriales antillaises ont déjà été rendues destinataires des préconisations de ce rapport

sont des établissements publics chargés d'une mission de régularisation foncière et non de protection de l'environnement. La mission de répression des atteintes à l'environnement est exercée, comme l'a indiqué M. le rapporteur, par le Conservatoire du littoral et l'Office national des forêts. Il faut donc veiller à ce que chaque

Dans certaines régions à vocation agricole, par exemple la Normandie, de multiples exploitations souterraines ont été ouvertes. Ces exploitations artisanales abandonnées, appelées marnières, peuvent, par dégradation naturelle sous l'effet des eaux d'infiltration, provoquer des effondrements de surface. Cet amendement vise à anticiper ce risque naturel important, complexe et difficile à traiter tant techniquement qu'administrativement. Le risque lié aux cavités souterraines reste, dans la plupart des cas, insoupçonnable jusqu'à ce que l'effondrement Cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle du code de l'environnement, qui a été modifié par l'article 224 de la loi de finances pour 2021. La suppression de la référence explicite aux marnières à l'article L. 561-1 du code de l'environnement constitue uniquement une simplification rédactionnelle et non une diminution du périmètre d'intervention du Fonds, ainsi que nous l'avions clarifié lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2021. Les effondrements de cavités souterraines et des marnières- il est vrai qu'en Normandie ces phénomènes sont particulièrement présents - sont une forme de mouvement de terrain. Cet amendement est donc pleinement satisfait. Au contraire, cet ajout pourrait avoir des effets indésirables sur d'autres textes. Indiquer que les effondrements de marnières

Compte tenu des spécificités des territoires ultramarins dans le champ de la gestion des règles de la loi Littoral, il convient que les collectivités locales concernées soient consultées sur les mesures d'adaptation pour la zone dite des cinquante pas géométriques. la ministre, vous avez indiqué en séance publique à l'Assemblée nationale que le Gouvernement prévoyait naturellement une concertation avec les collectivités territoriales et les parlementaires directement concernés par le projet d'ordonnance. Cet amendement a pour objet d'acter dans la loi le principe de cette concertation et les avis et recommandations des collectivités et parlementaires concernés. Cette consultation entre l'État et les collectivités

est à Mme la ministre. Cet amendement vise à inclure la mission d'adaptation des territoires au recul du trait de côte au sein de la compétence Gemapi. Pour favoriser la bonne coordination des actions en faveur de la prévention des inondations de la gestion des milieux aquatiques et de gestion du trait de côte, de gestion du trait de côte, cette mission est élargie aux actions d'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Dans cette perspective- c'est le point le plus important que je tiens ici à souligner les collectivités qui le souhaitent auront la possibilité d'utiliser la taxe Gemapi pour financer les opérations de recomposition spatiale. Ainsi, les collectivités disposeront d'une ressource fiscale dédiée pour engager leurs projets de recomposition des territoires, en plus des financements que j'ai déjà eu l'occasion de

Je rappelle que la Gemapi est une compétence obligatoire pour les communes ou les EPCI à fiscalité propre, selon les cas. Sous couvert de créer une nouvelle possibilité de financement, le Gouvernement propose en fait d'étendre le champ des compétences obligatoires du bloc communal. Il me semble que cette proposition conduit à acter le fait que la gestion du recul du trait de côte sera bel et bien, dans l'esprit du Gouvernement, une compétence locale et non une compétence partagée entre l'État et les collectivités. Cela revient clairement à opérer un transfert de responsabilité de l'État

Le rendement de la taxe Gemapi a atteint environ 200 millions d'euros en 2019. Plafonné à 40 euros par habitant, le rendement maximal de cette taxe pourrait atteindre 2,5 milliards d'euros à l'échelle nationale ; pour les seules communes littorales, ce chiffre ne dépasserait pas 250 millions d'euros. Or ce montant n'est jamais atteint et l'acceptabilité de telles hausses par le contribuable local est plus qu'incertaine, d'autant que cela ne permettrait pas de couvrir les dépenses liées au recul du trait de côte. Enfin, la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales a pour effet de réduire fortement l'assiette de la taxe

L'adaptation des territoires au recul du trait de côte, défini dans le projet de loi comme résultant soit de l'érosion côtière, soit de l'élévation permanente du niveau de la mer, devient donc une compétence des communes à l'échelon des EPCI. En creux, ainsi que le soulignent les associations, cette rédaction permet à l'État d'écarter l'idée d'une compétence partagée avec les collectivités. Il convient d'abord de rappeler que la taxe Gemapi est déjà insuffisante pour répondre à son périmètre initial. Le financement local de l'adaptation au recul du trait de côte par la taxe Gemapi pose donc des difficultés évidentes : l'échelle de solidarité fiscale est celle de l'EPCI, c'est-à-dire une échelle

de façon significative le nombre de redevables, puisque le périmètre ne comprend plus les foyers qui s'acquittaient auparavant de cette taxe. Ainsi, une hausse de la fiscalité Gemapi aura un effet concentré sur les propriétaires, les résidences secondaires et l'économie locale, ce qui pose la question de l'acceptabilité locale. Le rendement de la taxe ne permet pas du tout de couvrir l'intégralité des besoins cumulés- gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations et adaptation au recul du trait de côte. termes, cela revient à faire porter à l'échelon local la responsabilité politique et le poids financier de cette hausse de fiscalité sans pour autant répondre aux besoins qui concernent non seulement les logements, mais également les infrastructures, équipements et activités économiques liées. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet amendement.

2195. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

résultat du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,

La violence inouïe de l'ouragan Irma en 2017 est d'ores et déjà entrée dans l'histoire. Avec des vents qui ont effleuré les 300 kilomètres-heure, il s'agit du cyclone tropical le plus sévère observé aux Antilles. Les cyclones de ce type sont de plus en plus à redouter perspective, le présent amendement tend à créer une expérimentation pour cinq ans au titre de l'article 37-1 de la Constitution, limitée aux territoires ultramarins, d'un état de calamité naturelle exceptionnelle. Trois conditions cumulatives seront nécessaires pour y prétendre : un aléa naturel majeur, une atteinte au fonctionnement normal des institutions et un danger grave et imminent. imminent. Les conséquences de cette déclaration, la présomption d'urgence ou de force majeure qui s'y attache et les conditions de renouvellement de l'état de calamité naturelle exceptionnelle

de juillet 2019, après six mois de travaux, la rapporteure de cette mission, Nicole Bonnefoy, avait présenté son rapport. Le 27 novembre 2019, une proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles était déposée pour en

à l'ensemble des études et travaux de réduction de vulnérabilité pour les particuliers, et non plus seulement à ceux qui sont définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels. J'ajoute que le sujet a fait l'objet d'une question

du Gouvernement ? Le Gouvernement est déterminé à faire évoluer le régime des catastrophes naturelles pour permettre des indemnisations plus rapides et rétablir la confiance dans un régime qui a fait ses preuves mais qui manque parfois de transparence. C'est notamment l'objet de la mission d'inspection qui a été confiée au CGEDD et à l'IGF sur le retrait-gonflement des argiles.

des débats, le Gouvernement juge indispensable de traiter l'intégralité de la réforme des catastrophes naturelles dans un texte plutôt que par morceaux

au retrait-gonflement des argiles. Le rapport sera publié très prochainement. Cela permettra d'alimenter les travaux législatifs en cours pour améliorer les indemnisations de ces sinistres. Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques. J'indique par avance que, pour les mêmes raisons,

Afin de respecter ce principe, les communes vont devoir privilégier la densification des zones déjà urbanisées. Or, dans certains cas de figure, et en l'état de la législation, la densification est parfois rendue impossible. Par exemple, un immeuble ou une partie d'immeuble servant de local à vocation commerciale ou médicale et se trouvant en zone PPRI ne peut pas être destiné à de l'habitation. Même les locaux se situant aux étages supérieurs et ne présentant donc pas de risque imminent en cas d'inondation ne peuvent être changés de destination. Dans quelle mesure le changement de destination augmente-t-il la vulnérabilité dès lors que ces locaux sont au-dessus du niveau inondable ? Comment peut-on justifier qu'il n'y ait pas de risque pour les habitants actuels et interdire en même temps la transformation au même étage de locaux commerciaux en locaux d'habitation ? De surcroît, un tel changement de destination de commerce en habitation ne peut légalement se faire qu'à condition de prouver que, dans le passé, le local ou l'immeuble était à usage premier d'habitation. Le principe de vulnérabilité est abusivement évoqué dans les zones PPRI, même dans les derniers étages d'un immeuble. Nous sommes là dans l'incohérence de la loi et du règlement qui la traduit. L'objet du présent amendement est de clarifier l'application du principe de vulnérabilité à ce cas de transformation de local commercial en local d'habitation, sans accroître le risque pour l'habitant, tout en concourant à la densification nécessaire à l'atteinte du « zéro artificialisation nette L. 562-1 du code de l'environnement, en vertu duquel les PPRN peuvent délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles

et relève davantage d'une application statistique reposant sur quelques observations de niveaux d'eau atteints. Des centres-bourgs se retrouvent intégralement classés en zone rouge, à risque fort, c'est-à-dire inconstructibles et non aménageables. Ces classements accentuent le phénomène de désertification des zones rurales, des centres-bourgs et font obstacle à leur développement. Cela va par ailleurs à l'encontre des objectifs de sobriété foncière et de densification Cet amendement a donc pour objet de permettre, lors de l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation, la réalisation d'une évaluation des conséquences de l'application du plan envisagé sur l'attractivité économique des communes et le risque de désertification des centres-bourgs, afin de pouvoir, le cas échéant, ajuster les mesures du plan ou, mieux, les anticiper. Cet amendement se veut pédagogique vis-à-vis des services de l'État. Il s'agit d'améliorer la cartographie proposée et de mieux tenir compte de la réalité du terrain,

Gouvernement ? Je tiens à le souligner, un PPR a vocation non pas à figer un territoire, mais à lui permettre d'évoluer sous réserve d'une bonne prise en compte des risques et d'une réduction de sa vulnérabilité. Ainsi, même en zone d'aléas les constructions nouvelles sont autorisées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, sous réserve de réduire la vulnérabilité globale. Votre crainte de désertification n'est donc pas fondée, et les inondations fréquentes que l'on peut observer régulièrement soulignent l'impérieuse nécessité de tenir compte d'un tel phénomène dans l'aménagement du territoire. Les nombreux dégâts de l'automne dernier dans les vallées des Alpes-Maritimes ou voilà peu dans l'Aude nous le rappellent. En outre, le PPR n'est pas un outil adéquat pour effectuer une prospective économique de l'attractivité d'un de l'attractivité d'un territoire. Les enjeux socio-économiques du territoire sont toutefois pris en compte lors de l'élaboration du PPR à l'occasion des concertations avec les acteurs locaux, notamment les communes. Enfin, il n'y a aucune contradiction entre les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols

par la mise en place d'incitations fiscales pour les propriétaires, afin de réaliser les travaux renforçant la résilience de leurs bâtiments. Nous proposons de créer, sur le modèle du CITE, un crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement, afin d'améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles. Le taux de ce crédit d'impôt serait égal à 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 euros par personne à charge. Tel est l'objet du présent amendement.

suggéré de permettre de classer le phénomène d'échouages massifs d'algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle. En effet, le rapport interministériel analysant ce phénomène indique que la raison principale du refus de la commission de catastrophe naturelle de valider ce classement était l'impossibilité de pouvoir constater son caractère anormal faute de données de long terme. terme. Le fait qu'un phénomène soit inédit et peu étudié ne peut pas constituer un argument valide pour refuser de le considérer comme une catastrophe naturelle, à plus forte raison eu égard aux mutations de la planète du fait du réchauffement climatique. climatique. Cet amendement vise donc à remédier à un tel état ? Madame la sénatrice, vous avez raison, les sargasses posent de nombreuses difficultés aux territoires qui en subissent les échouages. Il y a d'abord des problèmes sanitaires potentiels relatifs aux émissions de gaz ; c'est du sulfure d'hydrogène. ensuite des difficultés économiques, car les sargasses nuisent au tourisme sur les littoraux et nécessitent des investissements massifs pour faire face aux échouages. Devant un tel constat, le plan Sargasses I a été mis en place par le Gouvernement dès l'année 2018. Il a d'ores et déjà permis de mettre en oeuvre des solutions de collecte

nous savons qu'il y a un vrai sujet à cet égard -et de débloquer des financements en matière de recherche et d'innovation, à hauteur de 8,5 millions d'euros. Le Gouvernement prépare actuellement le plan Sargasses II, qui fera l'objet d'une concertation courant de cette année. En revanche, les sargasses ne peuvent pas être considérées comme un risque naturel majeur et faire ainsi l'objet d'une introduction dans le régime « catastrophe naturelle », qui s'appuie sur des assurances auto et habitation. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

est à Mme la ministre. Cet amendement vise à instaurer un cadre législatif pour l'utilisation de drones par les agents concourant à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux. Les effets du dérèglement climatique se manifestent notamment par une évolution de l'érosion du trait de côte, mais aussi par des inondations en provenance de l'intérieur des terres. L'utilisation de drones offre donc une belle occasion de pouvoir mener correctement les travaux de cartographie du littoral, de disposer de meilleures connaissances des

dans un cadre rigoureux. C'est pourquoi le présent amendement vise à instaurer une information préalable du public lorsque les survols sont susceptibles de rendre possible l'identification des personnes physiques, à cantonner les destinataires des enregistrements aux personnels ayant besoin d'y avoir accès pour l'exercice de leur mission de connaissance et de prévision des phénomènes naturels dangereux et à limiter à six mois la conservation des enregistrements qui contiennent des données à caractère personnel. que seuls les agents habilités seront destinataires des enregistrements. Il s'agit également de prévoir l'information préalable du public concernant le survol d'une zone par un drone lorsque les prises de vue risquent de permettre l'identification de personnes physiques. De telles précisions permettent d'assurer un meilleur équilibre entre le renforcement de la connaissance scientifique sur l'évolution de certains phénomènes naturels